du piège du narcotrafic. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 4.

direction ou organisation de trafic de stupéfiants ; production illicite de stupéfiants en bande organisée ; importation et exportation illicite de stupéfiants en bande organisée. La lutte contre le blanchiment doit se fonder sur la diffusion et la mise en œuvre des compétences de l’État des enquêtes patrimoniales.

pour renforcer l’arsenal des moyens juridiques et opérationnels mis au service de la lutte contre le narcotrafic. Ce texte outille les services d’enquête, les magistrats et les auxiliaires de justice, ainsi que les maires, qui se trouvent en première ligne. Ces moyens doivent être efficaces, puissants et coordonnés,

sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée. Cette mesure est essentielle pour lutter contre le blanchiment d’argent et la pénétration de l’économie légale par des activités criminelles organisées. C’est en privant de manière systématique les organisations mafieuses de leurs profits illicites

Nous sommes convaincus que la saisie et la confiscation des produits d’infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance. Outre son caractère dissuasif, la peine de confiscation a une

Il a pour objet de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné sur le fondement de l’article 131 21 du code pénal. Un dispositif analogue est prévu à l’article 222 49 du même code, qui prévoit la confiscation obligatoire

Il s’agit d’agir vite, une procédure d’urgence, pour éviter la dissolution ou le transfert d’avoirs liés au narcotrafic à l’international. À la différence de la saisie ou de la confiscation, le gel ne signifie pas la prise de possession du bien par l’autorité judiciaire, mais seulement la possibilité d’en disposer.

Le gel administratif des avoirs se distingue ainsi clairement de la confiscation judiciaire, qui relève, quant à elle, d’une décision de justice entraînant la perte définitive de propriété.

la commission d’enquête ayant mis en lumière l’engorgement des prétoires et les longs délais d’audiencement. Il convient par conséquent d’outiller les magistrats, afin d’éviter la dissolution ou le transfert des avoirs à l’international durant des périodes susceptibles de s’étirer.

En outre, le recours direct au greffe de la chambre de l’instruction est peu courant, de sorte qu’un appel classique au greffe du tribunal judiciaire concerné apparaît plus approprié. Enfin, l’amendement a pour objet la possibilité pour le justiciable faisant l’objet de la saisie ou du gel des avoirs de solliciter du magistrat

M. Laurent Burgoa. Le présent amendement a pour objet de permettre aux procureurs de la République du parquet national anticriminalité organisée et à ceux des juridictions interrégionales spécialisées de transmettre des informations aux services de renseignement concernant les procédures portant sur des faits d’évasion en bande organisée. L’attaque d’Incarville a rappelé de manière dramatique les capacités dont disposent les délinquants particulièrement chevronnés pour s’extraire des mains de la justice. Par voie de conséquence, les services judiciaires et de renseignement doivent agir de concert en échangeant le maximum d’informations, afin d’éviter toute tentative d’évasion et d’atteinte à l’intégrité des agents et des bâtiments de l’administration pénitentiaire. L’extension du champ des procédures judiciaires dont les éléments peuvent faire l’objet d’une transmission aux services de renseignement, proposée opportunément par la commission des lois du Sénat, serait donc utilement complétée par cet amendement.

ces axes sont décrits dans l’article – analyse des informations, coordination des acteurs, participation à la stratégie et concours à la politique nationale

les contrôles ne sont pas aussi poussés qu’ils devraient l’être. À titre d’exemple, sur le port du Havre, 93,5 % des déclarations sont dédouanées en moins de cinq minutes,

parfois au détriment de la rapidité, et cela peut contribuer de manière décisive à la lutte contre le narcotrafic. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Cet article vise à expérimenter pendant deux ans le recours à la technique du renseignement algorithmique pour la détection des menaces liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tient à exprimer plusieurs réserves, eu égard à l’atteinte significative à la vie privée qu’implique la prolongation de cette expérimentation et, surtout, à l’opacité qui entoure ce dispositif. L’amendement du Gouvernement tend à supprimer les garde fous qui avaient été mis en place par les rapporteurs, en particulier l’obligation de transmission de l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

n° 70 rectifié . Le texte de la commission prévoit un mécanisme et un délai de judiciarisation dès lors que le renseignement recueilli par la technique de l’algorithme est de nature à caractériser la commission d’une infraction. Si la judiciarisation peut constituer objectif, le caractère obligatoire de la transmission au parquet risque d’interrompre l’action préalable des services de renseignement. Aussi cet amendement vise t il à supprimer ce caractère obligatoire, dans le respect du principe de séparation des moyens des services de renseignement et des services judiciaires. Une

sur l’expérimentation en cours, ses résultats et les contrôles qui seraient éventuellement nécessaires ! Il est pour le moins étrange de nous proposer de prolonger une expérimentation en nous demandant de faire confiance à son fonctionnement,

les groupes terroristes et, au delà, toutes les organisations criminelles tirent profit de la généralisation des messageries chiffrées et des difficultés qu’éprouvent les services de renseignement à accéder aux informations échangées sur ces plateformes. instaurer pour ces dernières une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires, afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et des données qui y transitent. Cet accès serait limité aux seules correspondances et données ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements, après avis de la CNCTR. Afin de garantir le respect de ces exigences de coopération, il est proposé de renforcer les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales

ce qui serait fait demain avec WhatsApp, Signal, Telegram ou d’autres applications. Actuellement, une grande partie, voire la totalité, des délinquants utilisent WhatsApp, Signal et Telegram, précisément

Notre collègue Cédric Perrin a raison : les technologies ont permis aux narcotrafiquants d’utiliser d’autres outils que leur simple téléphone.

donner les clés qui nous permettent de comprendre. Pensez vous un seul instant que les policiers et les gendarmes s’amusent à décrypter des conversations privées

C’est pourquoi nous tentons de mettre en œuvre de nouvelles dispositions. Sont elles perfectibles ? Probablement, et c’est tout l’intérêt de la navette parlementaire, mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments que vous nous

C’est ce critère qui distingue les deux infractions, qui ne se confondent pas, et j’imagine qu’un magistrat saura parfaitement faire la différence entre l’existence d’une préparation à une infraction et le fait de faire sciemment partie d’une organisation criminelle. Dès lors, comment définir une organisation criminelle ?

qui ne participent pas clairement à la préparation d’une infraction, mais qui participent très clairement à une organisation criminelle, et qui le savent. Soyons innovants si nous voulons gagner la lutte contre le narcotrafic.

de Muriel Jourda et de la commission des lois. Cet article reprend le modèle italien, qui a donné des résultats et dont nous avons souvent parlé depuis le début de la discussion. Il permet notamment d’étendre la caractérisation de la participation à l’association de malfaiteurs

pour appréhender pleinement les agissements des narcotrafiquants, en particulier de ceux qui agissent en haut du spectre, compte tenu de leur capacité à s’impliquer dans le trafic de stupéfiants tout en en restant suffisamment éloignés pour éviter une mise en cause judiciaire.

par des gens idéologiquement très éloignés de moi, qui lui reprochent son côté fourre tout. En tout état de cause, vous ne pouvez pas dire que la création de l’appartenance à une organisation criminelle de l’association de malfaiteurs. C’est un degré en dessous. Sur ce point là, vous ne m’avez pas convaincu. En revanche, je pense que la rédaction

Ils sous traitent et utilisent la main d’œuvre la moins chère possible, désœuvrée et si possible précaire. Si cet article va dans le bon sens, nous espérons que Pharos aura les moyens de traiter tous les signalements. Nous saluons l’ouverture de la réflexion sur la précarité des jeunes. Issus parfois

à mener toute activité ayant pour objet de faciliter le trafic. Cet amendement tend à protéger les mineurs. La commission d’enquête du Sénat sur l’impact

ces opérations de recrutement, constitue un élément de réponse nécessaire et bienvenu face à ce fléau abominable qui touche les mineurs. Tout autant que les autres sont exposés aux dangers du trafic, notamment à la violence des règlements de compte. Il est par conséquent légitime que le fait de les démarcher pour les recruter soit puni des mêmes peines.

En l’état du droit, l’article 132 4 du code pénal prévoit que, lorsque de telles infractions sont commises en concours, c’est à dire quand la seconde infraction a été commise avant qu’une condamnation n’ait été prononcée pour la première, les peines prononcées se cumulent entre entre elles, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Il en résulte un effet d’aubaine pour les narcotrafiquants, qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire, sans craindre, de fait, d’aggravation de la peine qu’ils encourent. du présent amendement constituent ainsi un élément de réponse face à la nécessité, soulignée avec force par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, de renforcer la lutte contre la poursuite des trafics en prison. De tels comportements, en effet, portent une atteinte grave à l’administration publique comme à l’autorité de la justice, atteinte dont la nature justifie déjà, en l’état du droit, une dérogation aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction pour les délits d’évasion ou de rébellion commise par un détenu. Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, cet amendement tend à cibler celle ci sur les infractions relevant de la criminalité organisée. Le cumul des peines encourues ne pourrait excéder un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Au surplus, la juridiction conserverait la possibilité, par décision spécialement motivée, de ne pas déroger aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction. Quel est l’avis de la commission ? Cet amendement

Les auteurs de l’amendement partent du constat que ces règles créent un effet d’aubaine pour les trafiquants, qui peuvent poursuivre leur trafic en prison sans risque de voir leur peine maximale aggravée. Ce constat est corroboré par des magistrats que nous avons auditionnés au cours de nos travaux et qui ont même plaidé pour la suppression pure et simple de ces règles de plafonnement des peines. Le ciblage proposé par les auteurs de l’amendement sur les infractions liées à la criminalité organisée nous paraît davantage proportionné et pertinent. Au demeurant, comme l’a rappelé notre collègue Burgoa, de telles dérogations existent déjà dans notre droit pour mieux réprimer des infractions qui défient l’autorité de la justice. Le passage par la prison est perçu par les narcotrafiquants comme une case à cocher dans leur cursus. Ils sont pleinement au fait des peines qu’ils encourent et du fonctionnement de notre justice pénale. Cette case prison, il nous appartient de la rendre plus dissuasive. Je sais que le garde des sceaux est déterminé à agir dans ce sens. La commission émet donc un avis favorable

Nous proposons également, en peine complémentaire, d’alourdir les sanctions pour les conducteurs.

cette mesure nous semble satisfaite par le droit existant. En effet, l’article 222 44 du code pénal permet déjà de condamner les personnes coupables des infractions liées au trafic de stupéfiants à la suspension de leur permis pour une durée de cinq ans, à l’annulation du permis avec une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans et à la confiscation d’un ou plusieurs véhicules.

la magistrature, « il est paradoxal d’envisager la prolongation d’une mesure de garde à vue pour répondre à une situation de danger imminent, alors que cette situation pourrait motiver la levée de la mesure pour incompatibilité médicale ». Il y a là une contradiction !

la personne placée en garde à vue continue de bénéficier des droits garantis par l’article 63 1 du code de procédure pénale, notamment celui d’être examinée par un médecin et assistée par un avocat, et ce chaque fois que la garde à vue sera prolongée.

que, entre la rédaction initiale de l’article et le dispositif que nous examinons ce soir, nous avons sensiblement renforcé l’encadrement de la mesure. Ainsi, nous en limitons la durée à cent vingt heures. Nous précisons les conditions dans lesquelles la prolongation exceptionnelle de la garde à vue peut être décidée, en prévoyant qu’un certificat médical, versé au dossier, établisse la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur son aptitude au maintien en garde à vue. Nous prévoyons des garanties pour la personne concernée à l’expiration de la quatre vingt seizième heure de garde à vue : la possibilité de s’entretenir avec un avocat ; le droit de demander un nouvel examen médical ; la possibilité de réitérer une demande tendant

des peines complémentaires applicables aux mules, en renforçant l’opérationnalité de la mesure et les garanties pour les personnes condamnées. La création de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans des aéroports et d’interdiction de vol a été recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France. Elle vise, pour protéger ces personnes,

En premier lieu, et à titre principal, il est indispensable de prévoir certaines garanties pour les personnes condamnées en ouvrant la voie, notamment pour faire face à une urgence médicale ou familiale, à une modification de l’application des interdictions de vol ou de paraître. Une telle décision de modification relèverait du juge de l’application des peines,

le même objectif paraît pouvoir être atteint de manière plus efficace par l’ajout d’un simple critère de conditionnalité, prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction de vol ou de paraître ne puisse être encourue que si l’infraction pour laquelle la personne est condamnée a été commise dans un aéroport ou un aéronef.

pour lutter contre le phénomène des mules. Le dispositif permettant au juge de l’application des peines de décider d’une modification de la peine vise à répondre à la préoccupation que vous aviez formulée, cher collègue, en commission. Des situations d’urgence médicale ou familiale, qu’il reviendra au juge d’apprécier, pourraient bien être prises en compte dans ces conditions. La commission émet donc un avis favorable

de constater que les ports n’étaient pas visés dans cet article. Si l’on considère qu’il faut empêcher les narcotrafiquants condamnés d’accéder à un certain nombre de lieux leur permettant

En premier lieu, il a pour objet d’étendre significativement le champ des contenus liés aux stupéfiants qui pourraient donner lieu à une demande de retrait, de déréférencement ou de blocage d’accès à internet par Pharos. Pour mémoire, l’article 12 vise précisément à étendre ce type de prérogatives aux contenus liés à l’offre et à la cession de stupéfiants,

Cette nécessité d’agir justifie bien à nos yeux une telle mesure, qui reste une atteinte importante au principe de liberté d’expression, puisque Pharos n’agirait ici que dans un cadre préventif de police administrative. Cela doit nous inviter à la prudence, si nous ne voulons pas fragiliser juridiquement ce dispositif utile et attendu et risquer

sont liés à la promotion de la consommation. Attention à ne pas faire disparaître d’internet la moitié du rap français, par inadvertance, au détour d’un amendement ! Nous n’ignorons évidemment pas que la lutte contre le narcotrafic est, aussi, un combat culturel et passe par un changement des mentalités vis à vis de la consommation. Cependant, la commission d’enquête ne s’est volontairement pas concentrée sur ces enjeux, qui appellent une analyse spécifique.

prépayées et de conserver ces informations pendant cinq ans pour les besoins de la lutte contre la criminalité organisée. Cette mesure correspond à la recommandation n° 19 de la commission d’enquête du Sénat. Les narcotrafiquants utilisent massivement des cartes SIM prépayées pour éviter toute identification et poursuivre leurs activités illégales de manière anonyme. Cet amendement vise donc à renforcer la traçabilité et l’efficacité des enquêtes pénales, tout en respectant le cadre juridique européen.

L’obligation de vérifier l’identité des acheteurs et de conserver ces informations pendant cinq ans constituera un outil précieux dans la lutte contre les trafics, sans pour autant violer les principes européens en matière de protection des données personnelles.

cela devient une condition pour obtenir des aveux et des preuves, dans un monde où l’on ne parle pas ou très peu,

Puisque la prison ne fait plus peur à une partie des narcotrafiquants, puisque les règlements de compte entre eux sont extrêmement violents, la prise de risque de quelqu’un qui se repentirait est énorme, pour lui et pour sa famille. C’est pourquoi

à l’établissement de la vérité et de coopérer. Il y a des mots pour désigner ces personnes.

ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d’exemption de peine prévues à l’article 132 78 du code pénal. Cela l’oblige à produire des éléments nouveaux pour pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice. telle situation constitue un lourd handicap pour cette personne, qui est ainsi pénalisée d’avoir révélé trop tôt des faits pourtant indispensables pour connaître l’étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle faisait partie. Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial que le coopérateur puisse avoir une visibilité et une garantie sur les conséquences de son engagement. Cela conditionne largement son adhésion au processus et la qualité des informations qu’il acceptera de divulguer. Cet abandonnement vise donc à corriger la situation

souhaitent apporter une précision bienvenue. Certes, la prise en compte des déclarations antérieures du repentir semble garantie par la compétence confiée au magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, mais il est sûrement plus clair de prévoir expressément que la décision du magistrat compétent peut se fonder sur les déclarations du prétendant au repentir antérieures à l’expression par celui ci de sa volonté de collaborer avec la justice. Toutefois, les amendements identiques n 115, 195 rectifié

en précisant que l’octroi du statut de collaborateur de justice s’effectuera en tenant compte des déclarations faites par la personne concernée avant que celle ci n’ait exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.

à la révélation du trafic par d’éventuels témoins, notamment en raison de l’ultraviolence des réseaux, qui suscite la peur des représailles envers les témoins et leurs proches. Afin de favoriser la protection des témoins menacés, le présent amendement ouvrir la possibilité de bénéficier, comme les policiers infiltrés et les repentis, de dispositifs dissimulant leur voix ou leur apparence physique et, d’autre part, à alourdir les peines encourues dans le cas où la révélation, directe ou indirecte, de l’identité d’un témoin protégé bénéficiant d’une identité d’emprunt s’est traduite par des violences à l’encontre de celui ci ou de ses proches, voire par la mort de l’une de ces personnes.

d’autoriser les enquêteurs et les magistrats, dans le cadre d’une instruction, à utiliser des techniques spéciales d’enquête qui permettent de recueillir des sons ou de prendre des images à distance. Aujourd’hui, les criminels savent protéger les lieux où ils exercent leurs activités. Ils en interdisent l’accès. Surtout, ils peuvent tendre des pièges aux policiers, et ceux ci, en voulant pénétrer dans ces lieux, se trouvent trouvent exposés à des risques majeurs. En tout cas, les criminels se protègent. Pour lutter contre un tel phénomène, il n’y a pas d’autre solution que de procéder à distance, avec des techniques spéciales, pour pénétrer des systèmes qui sont soit fixes, soit mobiles. Le Conseil constitutionnel avait considéré que donner trop de latitude pour pénétrer les systèmes mobiles, par exemple le téléphone portable, n’était pas suffisamment protecteur des libertés individuelles. Par cet amendement, nous ouvrons le champ de l’utilisation de ces techniques d’enquête. Pour les appareils fixes, nous mettons en place des dispositifs assez simples, à distance. Nous pouvons pénétrer un ordinateur. La procédure est relativement simple et légère.

d’abord, ce sont des décisions motivées, qui peuvent être soumises à recours. Ensuite, le champ d’intervention concerne les infractions les plus lourdes et les plus graves, du crime organisé, de la prostitution, des violences, des meurtres ou de la barbarie. Enfin, pour assurer ces protections, nous faisons en sorte qu’un certain nombre de lieux et de personnes soient protégés. Les lieux, ce sont des cabinets d’avocats, des cabinets de médecins, ainsi qu’un certain nombre de cénacles où il ne faut pas entrer trop facilement.